de l'Assemblée nationale. Il y a des raisons à cela, et vous les avez parfaitement explicitées. La définition des lanceurs d'alerte doit être claire, aussi claire que leur protection.

Avant même cette loi, les sénateurs centristes ont toujours été sensibles à cette question. Dès 2014, notre collègue Catherine Morin-Desailly, alors présidente de la commission de la culture, avait déposé une proposition de résolution visant à proclamer Edward Snowden citoyen d'honneur de la République française et à lui accorder l'asile politique. Moi-même, en 2015, j'avais proposé la création d'une commission d'enquête

apportée aux personnes qui fournissent une aide aux lanceurs d'alerte, appelées « facilitateurs ». Ces personnes jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'alerte. Il est donc essentiel de leur accorder une protection plus aboutie. aboutie. Le texte supprime également la hiérarchisation des canaux de signalement. Autrement dit, le signalement pourra désormais être effectué directement auprès d'une autorité externe et pas uniquement interne.

les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui portent sur un sujet d'une grande actualité concernant la protection des valeurs et des lois de la République : les lanceurs d'alerte. Ces derniers, en révélant certaines situations contraires à ces mêmes lois ou menaçant l'intérêt commun, peuvent en effet rendre d'importants services à notre société. est actuelle, cette question n'est évidemment pas entièrement nouvelle. Elle n'est pas étrangère au bien connu article 40 du code de procédure pénale, qui exige des agents publics qu'ils fassent part au procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont pu avoir connaissance. Il a toutefois fallu attendre 2016 et la loi Sapin II pour que l'on observe un véritable changement de paradigme et qu'émerge la première définition générale du lanceur d'alerte en France : le lanceur d'alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi » la violation d'une règle de droit, ou encore « une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Les lanceurs d'alerte bénéficient même d'une irresponsabilité pénale dans les cas où ils auraient porté atteinte à un secret protégé par la loi. Pour être considérés comme des lanceurs d'alerte et bénéficier de ce régime, ils doivent toutefois répondre à certaines conditions claires, en particulier de gravité des faits, et respecter certaines procédures. Le droit de l'Union européenne a, lui aussi, par la suite, consacré la protection des lanceurs d'alerte. La directive du 23 octobre 2019 concerne plus strictement la protection des lanceurs d'alerte portant sur des violations du droit de l'Union européenne. Elle est plus souple dans son application que la loi Sapin II, mais elle porte toutefois sur des domaines restreints. Ce faisant, elle aborde le lanceur d'alerte sous un prisme essentiellement professionnel. La proposition de loi déposée par nos collègues de l'Assemblée nationale a pour objet de transposer cette directive en droit français. Elle ne se borne toutefois pas à une simple transposition. Elle procède plutôt à une harmonisation des deux cadres juridiques, dans le but de renforcer les garanties globales dont bénéficient les lanceurs d'alerte. La commission des lois souscrit bien entendu à cet objectif. J'en profite pour saluer tout particulièrement notre rapporteur, Catherine Di Folco, qui a effectué un travail considérable sur le sujet et a encore permis la réalisation d'avancées depuis le dépôt du rapport, le mois dernier. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des mesures, pour certaines très techniques, qui ont été discutées en commission. Je remarquerai seulement que notre rapporteur s'est efforcé, par ses amendements initiaux, de garantir la cohérence de la transposition de la directive dans notre droit national. La directive et la loi Sapin II ne couvrent en effet en effet pas les mêmes champs : la directive européenne se concentre sur la violation des normes d'origine européenne, la loi Sapin II sur la protection de l'intérêt général et des lois de la République. La modification de la définition des lanceurs d'alerte en commission a cependant suscité un certain nombre d'inquiétudes. Celles-ci portent sur les effets que la nouvelle rédaction pourrait avoir sur les lanceurs d'alerte de bonne foi, ainsi que sur la complexité juridique qu'elle engendrerait. Afin d'apaiser ces craintes, et dans un souci de compromis, ce volet du texte pourrait donc évoluer au cours du débat : nous suivrons la position de notre rapporteur sur cette question. Le texte revient également sur les mesures de protection, dont l'amélioration doit permettre aux lanceurs d'alerte de ne pas craindre de représailles pour leurs actions. À des fins de clarification, il a été proposé de lister explicitement et d'un seul tenant les actions susceptibles de constituer des représailles. représailles. Par ailleurs, la commission a appelé de ses voeux la création d'un fonds de soutien aux lanceurs d'alerte, afin d'appuyer les mesures d'aide psychologique et financière prévues dans le texte. Corollaire de ces protections, le texte de la commission prévoit également des sanctions à l'encontre des lanceurs d'alerte de mauvaise foi. Ainsi, elle a réaffirmé que l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte n'a pas vocation à s'appliquer aux violations de domicile et autres accès frauduleux. La question des facilitateurs, ces personnes qui aident les lanceurs d'alerte dans leur démarche, a fait l'objet d'un débat en commission, pas tant sur son application aux personnes physiques que sur son application aux personnes morales. Cet aspect, étranger à la directive, n'est pas dénué d'intérêt, mais présente certains problèmes, qui ont conduit à la suppression de cette disposition, sur l'initiative de plusieurs de nos collègues. Bien entendu, ces personnes morales peuvent représenter un réseau de soutiens de bonne foi pour les lanceurs d'alerte, mais la rédaction du texte ne permettait pas de garantir que ce dispositif ne serait pas détourné de son objet et employé au service d'intérêts économiques ou politiques concurrents. Enfin, la proposition de loi organique aborde utilement le rôle du Défenseur des droits. La commission a voté les amendements du rapporteur prévoyant la nomination d'un adjoint du Défenseur des droits chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. d'alerte. Cet adjoint servira de cheville ouvrière au travail de qualification et d'accompagnement des lanceurs d'alerte et facilitera significativement le traitement des procédures de signalement externe. Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera ces deux textes dans la rédaction approuvée par la commission. je vous remercie

assez problématique, puisqu'elle revenait non seulement sur les avancées adoptées à l'Assemblée nationale, mais également sur certains des acquis de la loi Sapin II de 2016, qui protège aujourd'hui toute personne signalant ou révélant une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général.

En supprimant la notion d'intérêt général du cadre juridique des lanceurs d'alerte, la commission des lois du Sénat propose une définition régressive par rapport à celle de la loi Sapin II de 2016. Seul le signalement des crimes et délits sera ainsi envisageable, ce qui va à l'encontre des principes de la directive européenne relative à la protection des lanceurs d'alerte, laquelle prévoit clairement qu'aucun recul ne peut être accepté dans sa transposition en droit national. Très concrètement, si ce nouveau cadre venait à être adopté, un signalement comme celui qui a été effectué dans le cadre de l'affaire des ne serait plus possible. Je propose donc, par cet amendement, de rétablir une définition protectrice et inclusive du lanceur d'alerte comportant la notion d'intérêt général, tout en apportant deux modifications importantes. La première consiste à intégrer les personnes morales à but non lucratif dans cette définition. En effet, ces personnes sont des atouts essentiels pour l'information de nos concitoyens. Je pense Je pense par exemple aux associations de défense de l'environnement, que nous devons protéger. La seconde permettrait de renforcer le champ d'action de l'alerte en intégrant la divulgation relative à un risque sur la santé publique et l'environnement.

Comme l'a souligné l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2014, l'alerte doit permettre de couvrir l'ensemble des atteintes à l'intérêt général. Ainsi, doit être qualifiée de lanceur d'alerte toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu'elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé La suppression de la référence à la menace et au préjudice pour l'intérêt général aura un effet négatif majeur sur l'efficacité du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. À titre d'exemple, j'évoquerai le cas d'Irène Frachon.

Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de lanceur d'alerte. Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d'alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par ce statut. Or les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses. Par exemple, elles sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants, en vertu de l'article 121-2 du code pénal. Afin de redonner toute sa substance au texte proposé, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estime qu'il est nécessaire de revoir la définition retenue par la commission des lois, qui est contraire à l'esprit même de l'alerte. Nous vous proposons donc de rétablir la rédaction initiale de l'article 1.

J'avais regretté que notre commission des lois ait fait le choix de retenir une définition beaucoup trop restrictive. Je me réjouis donc du changement de position annoncé, qui devra néanmoins se confirmer.

et d'en faire un mécanisme pleinement démocratique, à rebours de certaines législations européennes, qui réduisent le mécanisme à une forme de « vigilantisme » exacerbé. Angèle Préville a d'ailleurs rappelé la position de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2014. Cette référence à l'intérêt général est également au coeur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, depuis 2008 et son arrêt, protège tous les lanceurs d'alerte signalant ou divulguant des faits contraires à l'intérêt général.

Dans le prolongement de ce qu'a dit Mme Goulet, je reconnais que Mme le rapporteur a fait un travail immense et a cherché à atteindre des équilibres sur la protection des lanceurs d'alerte. Néanmoins, la réécriture proposée de cet article 1 nous semble en retrait et pas totalement cohérente avec le droit européen- rappelons que cette proposition de loi vient transposer la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l'Union -, pas plus qu'avec le droit international. Il nous semble donc important de rétablir la rédaction initiale de l'article. Nous avons été ennuyés de constater la suppression des notions de menace et de préjudice pour l'intérêt général, remplacées par l'introduction d'un critère de gravité suffisante de la violation d'une règle

En distinguant le régime applicable selon que l'alerte porte ou non sur le champ de la directive et en supprimant la référence, pourtant en vigueur, aux menaces ou préjudices pour l'intérêt général, le texte de notre commission est revenu sur un apport important de la loi Sapin II, tout en introduisant une grande complexité pour tous les acteurs.

qu'il s'agisse des personnes à l'origine de l'alerte, bien sûr, mais également des entreprises, administrations et autorités chargées de la mise en oeuvre des canaux de signalement. La nécessité de revenir au texte de l'Assemblée nationale est assez largement admise, comme en témoigne la diversité des auteurs des amendements déposés en ce sens. Je pense bien sûr à l'amendement de notre rapporteure, que je salue, puisqu'elle a reconnu les écueils de la rédaction adoptée en commission. Il nous semble toutefois important et cohérent de tirer toutes les conséquences de ce rétablissement. J'y reviendrai lors de la discussion de l'article 3 s'agissant des conditions de divulgation publique. La parole

relevant du régime général de l'alerte. Je m'en expliquerai un peu plus longuement lorsque je donnerai l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements en discussion commune.

vise à reconnaître les personnes morales à but non lucratif, associations et organisations non gouvernementales, comme personnes morales pouvant bénéficier du statut de lanceur d'alerte. Comme je l'ai dit plus tôt ce matin, je pense qu'il faut rompre avec cette représentation des lanceurs d'alerte un peu romantique, comme étant des individus qui se lèvent seuls contre tous, face aux lobbies, et qui seraient les seuls à devoir être protégées. Donner l'alerte, c'est une responsabilité écrasante pour un individu seul. Les lanceurs d'alerte sont souvent isolés, en rupture avec leur hiérarchie, leur milieu social, dont ils cherchent à dénoncer les dérives. Un tel isolement, au-delà des angoisses et du malaise qu'il suscite, renforce l'omerta et le. Pour contrer cet isolement, les ONG et les associations jouent un rôle clé dans le processus d'alerte. Elles permettent aux lanceurs d'alerte de demeurer anonymes et de ne pas s'exposer, en relayant leur alerte en se faisant le porte-voix de leur dénonciation. Les lanceurs d'alerte doivent pouvoir être accompagnés juridiquement, psychologiquement, médiatiquement et socialement pour pouvoir surmonter l'épreuve qu'est le fait de donner l'alerte. C'est pourquoi nous proposons d'intégrer les personnes morales à but non lucratif dans la définition

entre les services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, mais aussi d'un consensus politique entre tous les groupes politiques du Parlement européen, y compris les conservateurs.

? Si elle est vraie, est-elle d'intérêt général ? Le reste concerne la morale, l'éthique, les situations privées individuelles, et cela ne doit pas regarder les juges, qui doivent uniquement trancher sur l'information elle-même.

est à Mme le rapporteur. Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il vise à clarifier la portée des exceptions liées à certains secrets protégés et à améliorer l'articulation du régime général d'alerte avec les régimes sectoriels.

pour présenter l'amendement n° 3. L'article 6 de la loi Sapin II, exclut du régime de protection des lanceurs d'alerte les faits « couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client L'article 1 de la présente proposition de loi ajoute le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et de l'instruction à cette liste. Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée « à l'exception des situations faisant l'objet de dérogations prévues par la loi Or, si des dispositifs d'alerte spéciaux existent en matière de secret-défense, de secret médical et de secret de l'avocat, aucun dispositif n'existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction.

Saisie d'une condamnation pour recel de violation de secret fiscal, la CEDH a estimé que la condamnation des journalistes concernés ne ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l'intérêt d'une société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.

la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte » n'est pas responsable pénalement.

La protection doit être générale et doit inclure les magistrats et les avocats. Notre droit protège déjà suffisamment le secret de l'instruction et de l'enquête. Un tel ajout est au mieux superfétatoire ; au pire, il sera utilisé abusivement contre le droit à lancer l'alerte.

L'article 6 de la loi Sapin II définit la notion de lanceur d'alerte et fixe les conditions de fond permettant de bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte. Ces conditions relatives à l'identité du lanceur d'alerte, à ses motivations, à la nature des informations révélées ou divulguées, à la manière dont le lanceur d'alerte en a eu connaissance et au degré de certitude que ces informations fournissent sur les violations visées. En ce qui concerne les motivations du lanceur d'alerte, notre commission a approuvé le choix fait par l'Assemblée nationale de supprimer le critère lié au caractère désintéressé de l'alerte, critère qui laisse une marge d'appréciation excessive au juge, ainsi que l'avaient souligné les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix dans leur rapport d'information. Note commission a également accepté que les informations révélées puissent fournir seulement des soupçons raisonnables qu'une violation a été commise, alors que le droit en vigueur exige que celle-ci soit manifeste. En revanche, notre commission a apporté deux modifications au texte de l'Assemblée nationale. En premier lieu, nous avons considéré que l'application du régime de protection, en particulier l'irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d'alerte qui portent atteinte à des secrets protégés ou violent une obligation de discrétion ou de confidentialité, ne se justifiait que si les faits signalés ou divulgués présentaient un degré de gravité suffisant. La commission a donc fait le choix de maintenir cette condition de gravité exigée par la loi Sapin II, sauf évidemment dans le champ matériel d'application de la directive ce choix était conforme à une recommandation du Conseil d'État, qui, dans son avis sur la proposition de loi, avait invité le législateur, avant de supprimer la condition tenant au caractère « grave et manifeste » des violations signalées ou d'introduire la référence à la notion « d'informations sur les violations » dans l'ensemble du champ couvert par les dispositions nationales, à évaluer l'impact de telles mesures, notamment en ce qui concerne les risques de détournement du dispositif de protection. En second lieu, alors que la loi Sapin II inclut dans le régime de l'alerte le signalement ou la divulgation de faits constitutifs d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général, notre commission s'est inspirée des termes de la directive en substituant à ces formules une référence aux actes ou omissions allant gravement à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. Sans emporter de conséquences majeures sur le fond, cette modification était motivée par le respect de la séparation des pouvoirs

Nous ne pouvons pas nous plaindre sans cesse d'une dérive vers le gouvernement des juges et laisser les tribunaux apprécier seuls, sans se référer aucunement à des règles de droit, les conditions dans lesquelles il est justifié de s'affranchir des règles communes, en particulier des secrets protégés par la loi ou des obligations légales de confidentialité.

mais la lutte contre l'évasion fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle, et la lutte contre l'optimisation fiscale est un objectif reconnu par le Conseil constitutionnel comme pouvant justifier des atteintes au principe d'égalité. Les révélations de M. Deltour auraient donc été couvertes par le régime de l'alerte tel que défini par la commission des lois. Quant à Irène Frachon, les faits qu'elle a eu le courage de révéler concernant la commercialisation du Mediator, dont les laboratoires Servier connaissaient les effets toxiques, ont été reconnus par le tribunal correctionnel de Paris comme constitutifs des délits de tromperie aggravée, d'homicide involontaire et de blessures involontaires. Il s'agit donc non pas seulement d'actes allant à l'encontre des objectifs fixés par la loi, mais d'actes illégaux, et même pénalement réprimés, qui entrent à ce titre pleinement dans le régime de l'alerte. J'espère que ces précisions auront dissipé vos

pour un lecteur non averti et, surtout, compliquer la tâche des organisations comme les administrations, les entreprises, etc., qui devront mettre en place des canaux de signalement interne et déterminer quels signalements entrent ou non dans le champ du régime légal de l'alerte. Je conçois en effet que cela puisse paraître complexe, et c'est pourquoi, afin d'apaiser les débats, je vous propose de revenir à la définition de la notion du lanceur d'alerte prévue par le texte de l'Assemblée nationale, tout en maintenant certains garde-fous

41 ont pour objet d'inclure parmi les lanceurs d'alerte des personnes morales à but non lucratif, ce qui ne me paraît pas du tout opportun. En effet, nous ne pouvons pas ignorer le risque que des associations de façade aux mains de puissances étrangères ou de puissances d'argent se constituent à seule fin de lancer des alertes tous azimuts pour déstabiliser les administrations et les entreprises françaises.

directe. Si la directive ne prévoit pas expressément un tel critère, elle exige néanmoins la bonne foi du lanceur d'alerte, ce qui serait incompatible avec la perception d'une rémunération. En second lieu, l'amendement vise à substituer à l'exigence de bonne foi une condition précisant que le lanceur d'alerte doit avoir des motifs raisonnables de croire que les faits qu'il signale sont véridiques au moment du signalement. est plus restrictive, car, en droit, la notion de bonne foi recouvre à la fois la croyance en la véracité de ce que l'on allègue et l'absence d'intention de nuire. Or les considérants de la directive font expressément référence à l'exigence de bonne foi. l'amendement n° 39, celui-ci deviendrait sans objet si l'amendement n° 94 de la commission était adopté. Enfin, les amendements n 3 et 40 visent à étendre le régime de protection des lanceurs d'alerte aux personnes qui porteraient atteinte au secret des délibérations judiciaires ou encore au secret de l'enquête et de l'instruction.

Dans la mesure où il existe des exceptions, légales ou jurisprudentielles, aux différents secrets visés ici, les divulgations qui entrent dans le champ de ces exceptions sont couvertes par le régime de l'alerte. La nouvelle rédaction du II du présent article proposée par la commission lève toute ambiguïté sur ce point.

Certaines associations et certains militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles- violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l'exercice de la liberté du travail -pour obtenir des images, des vidéos ou des amendement vise à soustraire ces informations du régime de l'alerte défini dans l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016. L'article 21 de la directive 2019/1937 exclut d'ailleurs les informations dont l'obtention ou l'accès constituent une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d'alerte.

Il s'agit de faire en sorte que le régime de protection des lanceurs d'alerte ne soit pas détourné de son objet par des personnes physiques ou des associations qui, au nom de l'intérêt général tel qu'elles le conçoivent, n'hésitent pas à faire intrusion dans des domiciles privés ou des locaux professionnels pour y prendre des documents ou y capturer des images dans le but de les diffuser sur internet. La commission, qui partage entièrement l'objectif visé, a retenu une solution différente, qui consiste, afin de lever l'ambiguïté du texte de l'Assemblée nationale, à écrire expressément dans la loi que l'irresponsabilité pénale dont bénéficient

soumis au secret de la défense nationale. Ainsi, un agent des services spécialisés de renseignement « qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du [code de la

Ils révélaient un scandale d'État concernant la vente d'armes et de technologies de surveillance à l'Égypte. En effet, l'exécutif savait que les armes et les technologies de surveillance utilisées par notre pays au nom de la lutte contre le terrorisme bafouaient les droits humains. La France s'est rendue complice de l'utilisation de ces renseignements par le régime égyptien pour traquer des trafiquants et des contrebandiers à la frontière avec la Libye. Cette affaire nous rappelle que le contrôle de l'action militaire de la France, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est un impératif démocratique. Avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a juridiquement encadré le statut du lanceur d'alerte dans le domaine de la défense nationale.

pas souhaitable d'affaiblir à ce point la protection de secrets nécessaires pour sauvegarder les intérêts supérieurs de la Nation. L'avis est défavorable sur ces trois amendements.

définis comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle ». La loi issue du vote de l'Assemblée nationale le 17 novembre 2021 étend également ce statut aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d'alerte. Il s'agit d'une avancée très importante, et vitale. Les ONG et syndicats jouent un rôle important afin d'aider les lanceurs d'alerte ou de lancer l'alerte en leur lieu et place pour leur permettre de rester anonymes, mais ils restent exposés juridiquement. Pour que ces personnes morales puissent continuer à assister les lanceurs d'alerte, une protection adéquate doit leur être accordée. En commission, la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d'alerte a

les dissuader de travailler avec les associations, ce qui est en contradiction avec l'esprit de la directive de 2019 qui vise à libérer la parole et à favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l'intérêt général. La parole

comment trouver le bon canal pour effectuer un signalement par exemple ? Quel cadre juridique faut-il respecter ? Ajoutons à ces interrogations les représailles, les conséquences financières, psychologiques et familiales qui pèsent sur les lanceurs d'alerte et entravent leur action. Surmonter ces difficultés relève de l'exploit. Il est donc nécessaire d'accorder aux syndicats et associations le statut de facilitateur, afin de leur permettre d'accompagner légalement une personne dans le processus de signalement, tout en leur garantissant une protection.

À l'inverse, en supprimant cette disposition, la commission des lois du Sénat s'incline devant la puissance des lobbys, soucieux de préserver les règles d'un capitalisme dominé par l'intérêt économique au détriment de notre intérêt général. En privant les syndicats et associations d'un tel cadre juridique et de son régime de protection, elle expose ces organisations aux représailles et aux menaces. Elle supprime une aide indispensable à celles et à ceux qui sont tentés de se lancer

car celle-ci répond à un objectif de protection de certaines catégories de personnes morales qui s'exposent en apportant aux lanceurs d'alerte une aide qui peut être déterminante. La version du texte proposée par nos collègues députés procède d'un équilibre qui a été largement soutenu,

Cette série d'amendements vise à accorder aux personnes morales à but non lucratif, à savoir notamment les associations et les syndicats, le statut protecteur de facilitateur,

Il me semble que le débat sur ce sujet s'est mal engagé et qu'il est devenu de fait assez confus. La portée de notre divergence avec l'Assemblée nationale ne doit pas être exagérée. Si une personne morale, telle qu'une association, assiste un lanceur d'alerte dans ses démarches, elle est protégée indirectement par les dispositions qui protègent le lanceur d'alerte lui-même, qu'elle bénéficie ou non du label de facilitateur. Je rappelle en effet que la protection des lanceurs d'alerte repose pour l'essentiel sur trois séries de dispositions : tout d'abord, une irresponsabilité pénale en cas d'atteinte à un secret protégé ensuite, une irresponsabilité civile dans le cas où, en signalant ou en divulguant des informations, le lanceur d'alerte aurait manqué à une obligation contractuelle de discrétion ou commis une faute ayant causé des dommages ; enfin, l'interdiction de certaines mesures de représailles. Sur le plan pénal, toute personne physique ou morale qui assiste un lanceur d'alerte ayant porté atteinte à un secret protégé pourrait être considéré comme un complice. Or, en l'application d'un principe général de droit pénal, il n'y a pas de complicité lorsque l'infraction principale n'est pas constituée. L'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte profite donc aux personnes qui l'assistent, qu'elles aient ou non le statut de facilitateur. Sur le plan civil maintenant, et plus particulièrement sur le plan de la responsabilité civile extracontractuelle, le même raisonnement doit être tenu. Il est irréaliste de penser qu'un tribunal puisse juger qu'une faute, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, a été commise du seul fait qu'il a aidé un lanceur d'alerte à accomplir les démarches que la loi autorise. Reste l'interdiction des mesures de représailles. Pour l'essentiel, les mesures de représailles interdites ne peuvent viser que des personnes physiques : une personne morale ne peut pas être licenciée, ni rétrogradée ou mutée. raison pour laquelle la directive du 23 octobre 2019 ne prévoit d'accorder le statut de facilitateur, qui permet donc de bénéficier de l'ensemble des protections offertes aux lanceurs d'alerte, qu'aux personnes physiques- vous l'avez vous-même rappelé en citant les termes Y ajouter les personnes morales ou certaines d'entre elles ne changerait pas grand-chose. Malgré tout, le débat a été brouillé par les inquiétudes suscitées par d'autres dispositions, en particulier la rédaction très extensive prévue par les députés concernant l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte et des facilitateurs. Des craintes très vives sont apparues quant au risque que le texte de l'Assemblée nationale puisse aboutir à protéger des associations qui sont aujourd'hui passibles de poursuites pénales en raison de leurs agissements, et qui doivent le rester, notamment lorsqu'elles violent des domiciles privés. C'est pourquoi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la commission a préféré revenir, à titre conservatoire, à une stricte transposition de la directive en réservant le statut de facilitateur aux seules personnes physiques.

se tourner vers des facilitateurs, ces associations très connues qui leur permettent d'être enfin entendus. Ces signaux d'alerte permettent d'avancer : il est par conséquent indispensable que des personnes morales puissent les accompagner et les soutenir.

de la commission ? La proposition de loi prévoit d'étendre le bénéfice des mesures de protection des lanceurs d'alerte « aux personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte,

de substituer à la notion de « personnes physiques » celle de « tiers », afin d'inclure les personnes morales. Ce dispositif est donc différent, puisqu'il accole le mot « tiers » à ceux de « personnes physiques ». Quoi qu'il en soit, je n'y suis pas favorable. Même si sa formulation n'est pas très explicite, la directive vise clairement les personnes physiques : elle cite l'exemple de collègues ou de proches de l'auteur du signalement, qui risquent de faire l'objet de mesures de représailles. Quel est l'avis du Gouvernement

Emboîtant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs du processus

la présente proposition de loi suivent cette évolution en créant, à l'article 5, une immunité pénale élargie pour les lanceurs d'alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d'alerte. Toutefois, cette protection n'est étendue qu'aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, et non à celles qui permettent aux lanceurs d'alerte de rester anonymes en relayant pour leur compte une alerte. Le présent amendement tend à remédier à cette situation en permettant à certaines catégories de facilitateurs de diffuser une alerte. Quel

En y réfléchissant, je me demande si ce n'était pas une fausse bonne idée. En cas de contentieux, la personne morale concernée serait contrainte pour établir sa qualité de facilitatrice et échapper à une condamnation de dévoiler l'identité du lanceur d'alerte, personne physique pour le compte de laquelle elle a agi. La protection de l'anonymat du lanceur d'alerte serait donc fragile et temporaire.

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile satisfait pour partie l'objet de cet amendement s'agissant de la défense de la liberté. Néanmoins, les refus répétés d'octroyer l'asile à Julian Assange ou à Edward Snowden

En réalité, ma chère collègue, sur le fond, vous avez satisfaction : si un lanceur d'alerte fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, il peut déjà se voir reconnaître la qualité de réfugié en France, soit sur le fondement de la Constitution, qui prévoit que la République peut donner asile à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, soit sur le fondement de la convention de Genève de 1951, qui prévoit l'octroi de la qualité de réfugié aux personnes persécutées pour des motifs politiques. Sur la forme, l'amendement pose aussi problème. Vous ne précisez pas quelle serait l'autorité qui serait habilitée à reconnaître à la personne concernée la qualité de lanceur d'alerte

-me semble à la fois peu pertinente et dangereuse. Peu pertinente, car la constitution de partie civile a pour objet d'obtenir du juge pénal la réparation des dommages matériels ou moraux causés aux victimes de l'infraction. Le lanceur d'alerte n'est pas toujours personnellement victime de l'infraction qu'il révèle. Il n'est pas non plus dépositaire des intérêts des victimes. Il n'aurait donc aucune réparation à obtenir en justice. Dangereuse, parce que l'objet réel de l'amendement est de permettre au lanceur d'alerte de mettre en mouvement l'action publique, alors même qu'il ne serait pas personnellement lésé par l'infraction. Autrement dit, c'est un moyen détourné d'introduire dans notre droit ce que l'on appelle « l'action populaire l'action populaire », c'est-à-dire la faculté pour toute personne de provoquer un procès pénal sur n'importe quels faits, en faisant fi des prérogatives du procureur de la République, auquel il appartient d'apprécier l'opportunité des poursuites. Pour ces raisons, l'avis est défavorable.

est à Mme le rapporteur. Cet amendement reprend une précision qui figurait dans le texte de l'Assemblée nationale. Les lanceurs d'alerte pourront désormais s'adresser directement à une autorité externe. Ils n'auront plus l'obligation d'effectuer d'abord un signalement en interne au sein de leur administration ou de leur entreprise. Néanmoins, selon la directive du 23 octobre 2019, les lanceurs d'alerte doivent être encouragés à emprunter prioritairement le canal de signalement interne, lorsqu'ils ne s'exposent à aucun risque de représailles et qu'il est possible de remédier efficacement à la violation constatée par cette voie.

est à Mme Mélanie Vogel. L'alerte ne devrait pas avoir de frontières, surtout quand elle concerne nos entreprises à l'étranger ou leurs sous-traitants. Nous le savons, les législations nationales dans le monde sont encore largement insuffisantes pour protéger les lanceurs d'alerte, surtout en dehors de l'Union européenne. En matière de protection de l'environnement, de défense des libertés ou d'évasion fiscale, les entreprises françaises doivent pouvoir être contrôlées quand elles sont présentes à l'étranger. Elles doivent être comptables des actions de leurs sous-traitants. Les faits de corruption pour remporter des marchés publics ou changer la réglementation nationale constituent l'un des enjeux majeurs de bonne gouvernance dans nombre de pays en développement. Ainsi, il nous paraît cohérent avec les objectifs du texte de protéger les lanceurs d'alerte quand ils, ou elles, travaillent directement ou indirectement pour une entreprise française établie à l'étranger. Une application restrictive de la loi risquerait, au contraire, de favoriser l'exportation de la corruption ou des atteintes à l'intérêt général en dehors des frontières nationales.

La question du champ d'application territorial de cette loi, et plus particulièrement des dispositions relatives au signalement interne, se pose effectivement. En principe, le droit français des sociétés s'applique aux sociétés dont le siège social est établi en France le droit du travail s'applique à tous les salariés travaillant habituellement en France, même si leur employeur est une société de droit étranger. Les dispositions ouvrant aux salariés le droit de procéder à un signalement interne et celles qui imposent à certaines sociétés de mettre en place une procédure spéciale de signalement interne peuvent se rattacher aussi bien au droit des sociétés qu'au droit du travail, si bien que l'on ne sait pas précisément quel est leur champ d'application. Le Gouvernement pourra sans doute nous éclairer sur le sujet Toujours est-il que l'amendement ne répond qu'imparfaitement à la question. En outre, qu'une procédure de signalement interne formalisée existe ou non dans la structure où travaille un salarié, le plus important est que celui-ci bénéficie des mesures de protection offertes par le régime lorsqu'il effectue un tel signalement interne. Or il n'y a là il n'y a là aucune ambiguïté. L'irresponsabilité pénale s'applique aux infractions susceptibles d'être poursuivies devant les juridictions françaises, en application des règles normales de compétence territoriale en matière pénale. En matière civile, l'irresponsabilité civile du lanceur d'alerte s'applique s'il a manqué à des obligations contractuelles découlant d'un contrat de droit français ou, en matière extracontractuelle et, en principe, si la faute a été commise en France.

doit même être encouragée « dans les cas de violations des droits de l'homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l'urgence d'informer le public impose de s'adresser directement à un journaliste ». L'alerte portée ainsi directement à la connaissance d'un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d'alerte qui effectue le signalement auprès d'une personne en position de la vérifier

je vous remercie

bat. Son affaire sera examinée par la Cour européenne des droits de l'homme le 2 février prochain. Il est question, ici, de liberté d'expression, à laquelle on oppose le secret des affaires, et ce même quand celles-ci sont illicites.

est à Mme le rapporteur. Cet amendement vise à apporter quelques précisions au contenu du décret qui devra réglementer la procédure de signalement interne.

pour les centres de gestion, possibilité utilement introduite en commission, de mettre à disposition de leurs communes membres et des établissements publics un dispositif mutualisé de recueil et de traitement des signalements. Nous proposons toutefois d'intégrer ce dispositif, allant dans le sens d'un allégement des collectivités territoriales, dans le code général de la fonction publique, afin de tirer les conséquences de l'ordonnance du 24 novembre dernier.

de mettre à disposition de l'ensemble de leurs communes membres, ainsi que des établissements publics du bloc communal, un dispositif mutualisé.

Or, dans sa réponse datée du 2 juin 2021, la Commission européenne considère que la directive impose à toute société employant plus de 50 salariés de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qu'elle fasse ou non partie d'un groupe, la mutualisation des moyens étant possible pour les seules sociétés comptant entre 50 et 249 salariés au sein d'un même groupe. En particulier, toujours d'après la Commission, la faculté laissée par la directive de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s'entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d'un même groupe. Il convient donc, pour éviter toute censure au regard des obligations de la directive du 23 octobre 2019, de supprimer les alinéas 23 à 27

à adapter, par voie réglementaire, les règles applicables en la matière aux spécificités des groupes de sociétés. Il s'agit d'exploiter toutes les souplesses prévues par la directive de 2019, afin d'éviter les redondances et de renforcer l'efficacité des procédures de traitement des signalements au sein des groupes. Il est en effet paradoxal de multiplier les canaux de signalement dans les sociétés d'un même groupe, alors que le pouvoir réel de décision est exercé par les dirigeants de la société mère, qu'eux seuls peuvent avoir une vue d'ensemble des dysfonctionnements du groupe et y remédier. C'est d'ailleurs pourquoi la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a imposé la mise en place d'une procédure spéciale de signalement au niveau de la société mère, et d'elle seule. Bien sûr, les lanceurs d'alerte doivent pouvoir s'adresser à un référent au sein de la société pour laquelle ils travaillent, si celle-ci atteint une certaine taille. Il ne s'agit pas de les obliger à saisir les instances de la société holding d'un groupe multinational, ayant son siège à New York ou à Singapour. L'objectif consiste, d'une part, à faire en sorte que l'information puisse remonter à la société mère si nécessaire et, d'autre part, à ne pas imposer de charges disproportionnées et inutiles aux sociétés de taille moyenne appartenant à un même groupe. Absolument rien dans le texte de la commission n'autorise ou n'oblige le Gouvernement à prendre des mesures qui iraient à l'encontre du droit européen. Bien au contraire, nous nous sommes inspirés de la doctrine que la Commission européenne a commencé à élaborer sur l'application de la directive, et nous avons souhaité laisser ouvertes laisser ouvertes toutes les portes qu'elle-même n'a pas fermées. La commission des lois est donc défavorable à l'ensemble des amendements tendant à supprimer les dispositions relatives aux groupes de sociétés introduites en commission, à savoir l'amendement n° 77

Seul le renforcement de l'indépendance des personnes gérant ces canaux paraît de nature à consolider la confiance des lanceurs d'alerte en la capacité de ces lignes internes à mettre effectivement un terme au problème dénoncé. Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé pour des salariés bénéficiant de mandats spécifiques, afin de leur permettre l'exercice de leurs fonctions en toute indépendance et sans crainte de représailles. Ainsi, le licenciement de ces salariés n'est possible qu'après une enquête de l'inspection du travail,

mener que le problème essentiel est la garantie d'un anonymat réel, souvent impossible, dans les faits, quand la plainte est traitée par la hiérarchie. Seul le renforcement de l'indépendance des personnes gérant ces canaux

Les amendements les désignent comme des « référents alerte », une expression absente du texte de la proposition de loi. En tant que salariés protégés, les référents alerte ne pourraient être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.

tout retrait du « mandat » de référent alerte. Dans ces mêmes amendements, il est précisé que le non-respect de cette procédure d'autorisation préalable serait constitutif du délit de représailles prévu à l'article 13 de la loi Sapin alors que ce délit concerne uniquement les représailles à l'encontre du lanceur d'alerte lui-même. Il y a donc là une incohérence, qu'il faudrait corriger. Sur le principe, je ne suis pas convaincue qu'il soit nécessaire d'accorder un statut aussi protecteur aux personnes qui seront chargées de recueillir et de traiter les signalements internes. Elles n'auront effectivement aucun pouvoir pour prendre des mesures correctrices dont les dirigeants de l'entreprise ne voudraient pas. Je ne vois donc pas comment elles pourraient se heurter à l'hostilité de leur employeur, au point d'être licenciées ou même mutées abusivement. Je note d'ailleurs que le référent « harcèlement sexuel », obligatoirement désigné dans les plus grandes entreprises, ne bénéficie pas en cette qualité du statut de salarié protégé. De même, le référent déontologue dans la fonction publique n'est pas spécifiquement protégé. Cela dit, nos collègues soulèvent effectivement la question des garanties d'impartialité et d'indépendance du traitement interne des signalements, garanties qui, selon la proposition de loi, devront être fixées par voie réglementaire. Je souhaite donc que le Gouvernement nous éclaire sur le sujet. Quel est

financiers clandestins). Entre-temps, M. Forissier a été licencié en octobre 2009 pour « avoir dénoncé de manière mensongère et réitérée l'existence d'un système de fraude fiscale et de comptabilité parallèle ». Tous ces faits ont été reconnus par la justice et la banque a été condamnée

Nous proposons ainsi de réunifier le régime de divulgation publique, que l'alerte s'inscrive dans le champ de la directive ou non. Tout d'abord, dans la rédaction proposée par nos soins, la divulgation publique reste soumise à des conditions exigeantes, et nous soutenons bien sûr cette nécessité d'équilibre. Ensuite, les arguments avancés par Mme la rapporteure pour rétablir la définition des lanceurs d'alerte s'appliquent ici pleinement. Distinguer le régime applicable selon le champ d'alerte apparaît comme une source de complexité et nuit à la lisibilité du dispositif global, que le présent texte cherche pourtant à affermir. Nous comprenons donc mal le choix de Mme la rapporteure de maintenir ce dualisme pour la divulgation publique, mais également d'intégrer un nouveau critère de gravité lorsque celle-ci n'entre pas dans le champ de la directive. Nous vous proposons donc, mes chers collègues, en cohérence avec le vote ayant eu lieu à l'article 1, d'adopter notre amendement tendant à rétablir, ici aussi, la version de l'Assemblée nationale. Les

alors que la précédente version prévoyait qu'une telle possibilité était ouverte « en cas de danger imminent ou manifeste ». Or il s'agit d'une atteinte à l'esprit de la directive, qui prévoit, en son article 15, que le danger en cause doit être imminent ou manifeste, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs. Au cours de la cinquième réunion du groupe d'experts de la Commission sur la directive de 2019, qui s'est tenue le 14 juin 2021, il a été souligné qu'une « loi de transposition qui ne reprendrait pas les conditions prévues à l'article 15 ne procéderait pas à une transposition correcte de la directive les conditions prévues par l'article 15 visent à trouver un équilibre adéquat entre l'intérêt public à mettre en lumière des fautes susceptibles de porter atteinte à l'intérêt public, d'une part, et à protéger les intérêts des personnes visées par l'alerte, d'autre part En application de l'article 25, qui prévoit que « la mise en oeuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive », cette possibilité de saisir la presse doit être maintenue pour l'ensemble des lanceurs d'alerte. En effet, dans le cas contraire, il s'agirait d'une régression du droit d'alerter le public puisque, en l'état actuel du droit, l'article 8 de la loi Sapin II prévoit une possibilité de saisir la presse en premier lieu en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, ce qui est plus large que la notion de danger imminent et manifeste.

alors que la précédente version l'autorisait. La position du Sénat serait de considérer que seul un danger manifeste, imminent et d'une gravité suffisante- ces trois conditions étant cumulatives -peut justifier de court-circuiter les procédures normales de signalement.

Cette série d'amendements porte sur les conditions dans lesquelles un lanceur d'alerte peut divulguer les informations dont il dispose, par exemple en les livrant à un journaliste ou en les publiant sur des réseaux sociaux. La proposition de loi prévoit de faire bénéficier de l'ensemble des mesures de protection prévues par la loi Sapin II, en particulier l'irresponsabilité pénale en cas d'atteinte à un secret protégé et l'irresponsabilité civile en cas de préjudice causé à autrui, le lanceur d'alerte qui divulgue ces informations, dans plusieurs cas de figure. Le premier cas est celui où le lanceur d'alerte a préalablement signalé les faits à l'autorité compétente et où celle-ci ne lui a pas apporté une réponse appropriée dans le délai imparti. C'est évidemment légitime. Il appartiendra au juge, le cas échéant, de dire si la réponse a été ou non appropriée. La commission des lois n'a donc rien changé à ce premier cas. Le deuxième cas est celui où le signalement des faits à l'autorité compétente soit ferait courir au lanceur d'alerte un risque de représailles, soit ne pourrait aboutir à aucun résultat. La proposition de loi mentionne par exemple l'hypothèse où des preuves peuvent être dissimulées ou détruites pendant le traitement du signalement par l'autorité compétente, mais aussi l'hypothèse où l'autorité est en situation de collusion avec l'auteur des faits. Là encore, la commission a maintenu le texte tel quel. Le troisième cas prévu par les députés, qui se sont alignés sur le texte de la directive, est celui où il existe un « danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ». Cette formulation n'est pas forcément n'est pas forcément très limpide ... Pour sa part, la commission a estimé que, dans le cas où le lanceur d'alerte ne s'expose à aucun risque de représailles en saisissant l'autorité externe, où aucune preuve ne peut être détruite et où il n'y a aucune raison de penser que l'autorité externe est en collusion avec l'auteur des faits, rien ne justifiait de court-circuiter la procédure normale de signalement externe et de rendre les faits publics, à moins qu'ils ne soient suffisamment graves et qu'il existe un danger à la fois imminent et manifeste. Cela me paraît parfaitement raisonnable et je voudrais prendre un exemple concret pour essayer de vous en convaincre. cas d'une commune où un permis de construire doit être délivré pour la construction de logements sociaux sur un terrain jusque-là non artificialisé. Un fonctionnaire de cette commune a de bonnes raisons de penser que les autorités municipales, vu l'urgence qu'il y a à construire de nouveaux logements sociaux, ont passé sous silence le risque que le projet ne perturbe gravement l'habitat d'une espèce animale rare, par exemple une espèce d'oiseau. Des irrégularités ont été commises et il existe un risque pour la protection de la biodiversité. Au vu des informations dont dispose le fonctionnaire, ce danger peut être considéré comme suffisamment grave et manifeste, sans pour autant être imminent, les travaux ne devant pas commencer avant un certain délai, un an par exemple. Quelle est la bonne méthode dans une société démocratique pour parer à ce danger ? Supposons que l'autorité externe compétente pour traiter ce genre de signalement soit le préfet. Le fonctionnaire peut également saisir le procureur de la République si des infractions pénales ont été commises ; il en a même l'obligation s'il s'agit de crimes ou de délits. Rien ne laisse penser que le préfet ou le procureur a un intérêt personnel dans l'affaire, que le fonctionnaire s'expose à des représailles en le saisissant, ni même que des preuves puissent être détruites. Selon moi, la bonne méthode consiste pour ce fonctionnaire à saisir le préfet ou, le cas échéant, le procureur, l'un et l'autre ayant les moyens de procéder aux investigations complémentaires nécessaires et, le cas échéant, d'empêcher que le projet ne voie le jour. Supposons que le Supposons que le préfet ou le procureur n'apporte aucune réponse au lanceur d'alerte dans le délai de trois mois. Alors celui-ci pourra révéler les faits à qui bon lui semble. Mais, selon moi, il n'y a, dans un tel cas de figure, aucune raison de se dispenser de la saisine préalable de l'autorité externe. Étendre trop facilement l'application du régime de protection des lanceurs d'alerte à des personnes qui s'affranchissent sans nécessité des obligations de confidentialité auxquelles elles sont soumises, voire des secrets protégés par la loi, c'est affaiblir inutilement ces obligations et ces secrets qui ont été institués pour de bonnes raisons. En l'occurrence, les fonctionnaires, comme les salariés de droit privé, sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle, qui est un corollaire de leurs obligations de loyauté vis-à-vis de leur employeur et qui contribue au bon fonctionnement des administrations et des entreprises et à la confiance qui doit régner en leur sein. Cette obligation de discrétion doit céder à des motifs plus importants comme la prévention d'atteintes graves à l'environnement, mais elle doit demeurer dans tous les cas où il n'est pas nécessaire de l'écarter.

Dans son souci de compromis, la commission a proposé à l'article 1- ce que le Sénat a accepté -de revenir à une définition unifiée des informations relevant du régime de l'alerte, en supprimant toute condition liée à la gravité des faits signalés ou divulgués, même lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la directive du 23 octobre 2019. En revanche, elle En revanche, elle entend maintenir ce critère de gravité lorsqu'il s'agit d'autoriser la divulgation publique directe des informations sans signalement préalable à l'autorité compétente. L'amendement n° 100 prévoit que, lorsque la divulgation publique d'informations « porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale », le régime de protection de la loi Sapin II ne s'applique que si le lanceur d'alerte a préalablement signalé les faits à l'autorité compétente, sans obtenir de réponse appropriée dans le délai. les cas de divulgation publique directe d'informations sans signalement préalable seraient exclus en cas d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. Cette exception s'impose à nous, en vertu de l'exigence constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle est également conforme à la directive, qui prévoit que les règles qu'elle édicte n'affectent pas la responsabilité qu'ont les États membres d'assurer la sécurité nationale ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. Quel est l'avis du Gouvernement ? Dans la

Le scrutin est ouvert.

le grand public a, par définition, intérêt à la connaître et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée « dans les cas de violations des droits de l'homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l'urgence d'informer le public impose de s'adresser directement à un journaliste ». L'alerte portée ainsi directement à la connaissance d'un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d'alerte qui effectue le signalement auprès d'une personne en position de la vérifier et de l'anonymiser par exemple. exemple. Quel est l'avis de la commission ? En premier lieu, cet amendement prévoit d'instituer de nouveaux cas où le régime de protection bénéficierait aux personnes ayant divulgué des informations, même secrètes ou confidentielles, sans les avoir préalablement signalées à l'autorité compétente, « dans les cas de violations des droits de l'homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l'urgence d'informer le public impose de s'adresser directement à un journaliste ». Cela n'ajoute en réalité pas grand-chose sur le fond, puisque la divulgation publique directe des informations serait permise en cas de danger grave, imminent et manifeste- nous venons d'en voter Sur la forme, il me paraît gênant d'introduire les notions de droits de l'homme et de libertés fondamentales sans les définir, ne serait-ce que par référence à des textes comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

de la commission ? La directive du 23 octobre 2019 protège strictement la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement. Elle prévoit que tout élément permettant d'identifier l'auteur d'un signalement ne peut être révélé qu'avec le consentement de celui-ci ou « lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l'Union ou le droit national dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités nationales ou dans le cas de procédures judiciaires [ ...] ». Or le texte de l'Assemblée nationale autorisait la divulgation de l'identité de l'auteur du signalement à l'autorité judiciaire sans autre condition.

chargée de signaler les atteintes à la santé publique et à l'environnement. Son rôle d'alerte recouvre plusieurs types de signalement : dénonciation d'activités illégales ou illicites, émission de signaux sur un danger ou sur un risque méconnu ou sous-estimé. Le principe de précaution est encore trop souvent ignoré quand il s'agit de protection de la santé de nos concitoyens ou de l'environnement. Par exemple, l'exposition des populations à certaines substances de la pétrochimie a un impact direct sur la fertilité des individus et les pouvoirs publics réagissent souvent trop tard. de régulation de nombreuses activités sont détournées par des secteurs économiques qui investissent la recherche et la production d'expertises pour amoindrir les preuves d'une éventuelle atteinte à la santé ou à l'environnement.

recouvre plusieurs types de signalements : la dénonciation d'activités illégales ou illicites et l'émission de signaux sur un danger ou un risque méconnu ou sous-estimé- souvent appelés « signaux faibles » -, qui nécessitent, le cas échéant, de prendre des mesures visant à en limiter les conséquences potentielles sans attendre d'avoir des certitudes,

de la commission ? Ces amendements, qui visent à élargir les attributions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, nous semblent largement satisfaits par le droit en vigueur, puisque cette commission est déjà compétente pour émettre les recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement. Les amendements mentionnent par ailleurs la faculté pour elle d'entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la santé et de l'environnement. Je ne suis pas certaine de comprendre la portée de cet ajout. La CNDASPE peut entendre qui elle souhaite et n'est obligée de révéler l'identité d'aucun de ses interlocuteurs. En revanche, elle n'a effectivement pas le pouvoir de contraindre des personnes à effectuer devant elle une déposition, ce qui est bien normal pour une commission administrative.

Enfin, il n'est pas opportun d'inscrire dans la loi de 2013 que la commission traite des alertes qui lui sont transmises en matière de santé et d'environnement, en application de la loi Sapin II. Précédemment, lors de l'examen de l'article 3, nous avons décidé d'habiliter le Gouvernement à désigner lui-même les autorités externes compétentes en fonction des matières. Laissons-lui la souplesse nécessaire : la CNDASPE n'a pas nécessairement vocation à se voir attribuer compétence pour traiter seule de toutes les alertes relatives à la santé ou à l'environnement, ce qui constituerait une charge de travail impossible à absorber. Avis défavorable sur les deux amendements.

part, de l'infraction de dénonciation calomnieuse, visée à l'article 226-10 du code pénal, qui permet de sanctionner « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ». Il s'agit, d'autre part, de l'infraction de diffamation prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui permet de sanctionner « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Quel est l'avis de la commission de la commission ? La directive prévoit « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations Or le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si les faits dénoncés sont passibles de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et si le destinataire est lui-même investi d'un pouvoir de sanction ou peut saisir l'autorité compétente. Compte tenu du large champ de l'alerte en droit français et de la nature des autorités externes qui sont désignées par décret, cette incrimination pénale ne couvre pas l'ensemble des signalements effectués de mauvaise foi. C'est ce qui justifie l'insertion de cet article. Avis défavorable

aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation. Toutefois, l'articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d'État est problématique. En effet, la jurisprudence administrative la plus récente confirme la sévérité la sévérité du juge administratif à l'égard des agents ébruitant les dissensions internes à l'administration : elle valide généralement les sanctions infligées à l'encontre des agents qui dégradent l'image des services administratifs.

De même, a été jugée légale la sanction infligée à un fonctionnaire du service de santé des armées ayant écrit un livre et participé, sans autorisation de sa hiérarchie, à des émissions de télévision pour dénoncer des dysfonctionnements qu'il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal. La rigueur de l'obligation de réserve semble ainsi exposer les agents publics lanceurs d'alerte à des sanctions quasi systématiques dès lors qu'ils s'expriment publiquement, d'autant que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg rejoint largement celle du juge français sur ce point

pour l'obtention du statut de lanceur d'alerte sont remplies.

La discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes par rapport à d'autres pour des motifs prohibés, comme le fait d'avoir lancé l'alerte, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour atteindre ce but ne soient appropriés et nécessaires. La suppression de la possibilité de reconnaître ce type de discrimination contre les lanceurs d'alerte crée une grave rupture d'égalité entre entre lanceurs d'alerte et salariés discriminés pour d'autres motifs. Or une telle différence de traitement ne peut être objectivement justifiée, comme l'exige la jurisprudence du Conseil constitutionnel. De plus, cette suppression peut encourager les employeurs à mettre en oeuvre des mécanismes de discrimination inédits pour éviter des censures de la part des conseils de prud'hommes. Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposent de rétablir le champ initial de protection. Ils veulent ainsi permettre aux juges de reconnaître l'existence de discriminations indirectes contre les lanceurs d'alerte.

Sur la forme, il me semble essentiel que l'ensemble de ces mesures soient réunies dans une seule disposition : la multiplicité des renvois nuit à la lisibilité du régime et pourrait dissuader certaines personnes de lancer une alerte, faute de vision claire quant aux protections qui leur seraient accordées.

C'est le cas des travailleurs indépendants, notamment des travailleurs des plateformes, ainsi que des agents publics soumis à un statut particulier- on pourrait citer d'autres exemples encore. Pourtant, ces personnes sont tout aussi susceptibles de lancer une alerte que des salariés ou des agents publics relevant du statut adopter la rédaction du Gouvernement, c'est se résoudre à laisser certains lanceurs d'alerte sans protection contre d'éventuelles représailles. Je vous propose donc de vous en tenir au choix de la commission, qui comble ces lacunes et qui est guidé par la volonté de protéger tous les lanceurs d'alerte, quelle que soit leur catégorie professionnelle. concerne les amendements identiques n 11 et 50, je précise que le devoir de réserve impose uniquement aux agents publics de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression. ne sont en aucun cas incompatibles avec le fait de lancer une alerte. Surtout, comme tout citoyen, les agents publics bénéficient des protections prévues par cette proposition de loi. Une sanction injustifiée, fondée sur la méconnaissance du devoir de réserve, aurait le caractère de représailles et serait, de fait, illégale. Enfin, l'amendement n° 59 tend à préciser que les représailles peuvent être directes ou indirectes. Pour des raisons de clarté, la commission a fait le choix de coller à la terminologie de la directive, laquelle n'établit pas de distinction selon la nature des représailles. Quoi qu'il en soit, la liste des mesures prohibées me paraît suffisamment détaillée et explicite. Il ne fait aucun doute qu'elle recouvre les discriminations directes et indirectes. À mon sens, cet amendement est satisfait. En résumé, la commission est défavorable aux amendements n 84, 11, 50 et 59.

ou Slapp (pour, désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d'alerte, un détracteur ou un opposant afin, non pas de le faire condamner, mais de le faire taire en l'épuisant financièrement, moralement et nerveusement. Ces poursuites présentent un certain nombre de caractéristiques communes désormais connues- nous en avons plusieurs exemples.

un lanceur d'alerte pourrait donc être contraint à la rembourser. Avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête, aucun lanceur d'alerte ne se risquera à demander le bénéfice d'une telle provision.

puisse décider, pour des considérations d'équité, que la provision versée reste définitivement acquise au lanceur d'alerte dans le cas où celui-ci serait la partie perdante

envers un lanceur d'alerte. Le texte de l'Assemblée nationale ne permettait pas à l'auteur d'une mesure dont le caractère de représailles est en cause de se défendre sur le fondement d'une méconnaissance de la procédure d'alerte. Or, si le droit d'alerte est encadré, c'est pour assurer un équilibre avec la protection d'autres intérêts également légitimes. Des sanctions peuvent se justifier lorsque ces intérêts ont subi des atteintes en dehors du cadre légal.

à l'aide de tout type de magnétophone, constitue un procédé susceptible de porter atteinte à l'intimité de la vie privée. Or, dans l'hypothèse de malversations ayant lieu au sein des entreprises, procède régulièrement à des enregistrements pour accumuler des preuves de l'alerte. Ces preuves sont recevables devant les juridictions pénales afin de qualifier un délit ; elles sont fréquemment utilisées en matière de délits financiers et de corruption. Il nous paraît donc indispensable de faire confiance à la sagesse des juridictions pour déterminer, en chaque espèce et dans le cadre bien balisé du droit au procès équitable, si l'atteinte à la vie privée était nécessaire au regard de l'atteinte portée aux intérêts des parties adverses. Voilà pourquoi nous proposons de rétablir cet article dans la version

l'avis de la commission ? Ces quatre amendements

En l'état, le code pénal protège les lanceurs d'alerte contre les poursuites pénales à raison des atteintes à un secret protégé par la loi, dès lors qu'ils ont respecté les conditions légales de fond et de forme de l'alerte.

? d'un abus de confiance ? de l'intrusion dans un réseau informatique, pour y récupérer des informations afin de les diffuser ? de l'intrusion dans une propriété privée ? Ces ambiguïtés ont suscité de fortes inquiétudes, en particulier dans le monde agricole- je n'y reviens pas. Quoi qu'il en soit, la protection des lanceurs d'alerte n'autorise pas tout : ce n'est pas la loi de la jungle

la fin ne justifie pas tous les moyens. Dans un esprit de compromis, la commission n'est pas revenue sur le terme « soustraire ». En revanche, elle a tenu à inscrire expressément dans le présent texte que l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte ne s'étend ni aux atteintes à la vie privée ni aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Cette rédaction n'est pas des plus simples, mais elle a le mérite de lever toute ambiguïté.

il précise toutefois que cette irresponsabilité ne jouerait que dans le cas où le lanceur d'alerte aurait eu accès auxdites informations de manière licite. L'intention me paraît claire : dès lors qu'une personne violerait un secret protégé en divulguant des informations obtenues de manière illicite, par exemple au moyen d'une intrusion dans une propriété privée ou dans un système informatique, ou par un simple vol de document, elle ne bénéficierait d'aucune irresponsabilité pénale. C'est seulement si la personne avait accès licitement à ces informations qu'elle serait couverte.

fait de ce dernier un usage différent de celui pour lequel il lui avait été remis, ce qui pourrait être qualifié d'abus de confiance. Au bénéfice

Les personnes morales, en particulier les associations de la loi de 1901, jouent un rôle clé dans le processus d'alerte en relayant les alertes des lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de lanceur d'alerte. Il en va ainsi, par exemple, de l'association Greenpeace

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d'alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or les représailles dont elles peuvent faire l'objet sont nombreuses. En effet, En effet, depuis la réforme du code pénal de 1994, elles sont responsables pénalement des actes de leurs représentants. Qu'il s'agisse des incriminations de vol d'informations, de recel de secrets professionnels ou encore d'intrusion dans un système informatique, les dispositions pénales susceptibles d'être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d'alerte sont nombreuses. Or des poursuites engagées sur ces fondements donnent aux personnes visées par l'alerte la possibilité de demander au juge des actes d'enquête- perquisitions, saisies informatiques -de nature à permettre d'identifier la source d'une alerte relayée par une association. De telles poursuites compromettent donc la capacité des organisations en cause de protéger l'anonymat de leurs sources et, ce faisant, exposent les lanceurs d'alerte à des mesures ultérieures de rétorsion. Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d'alerte, mais risque de les dissuader de travailler avec des associations, en contradiction avec l'esprit de la directive européenne de 2019 qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l'intérêt général. Cet état de fait est en outre contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que la fonction « chien de garde », qui consiste à provoquer un débat public et à y contribuer, n'est pas l'apanage des journalistes professionnels,

l'avis de la commission ? Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a entendu réserver le statut de facilitateur aux seules personnes physiques. Quoi qu'il en soit, le secret des sources ne me paraît tout simplement pas transposable au cas des lanceurs d'alerte. Il a été conçu spécifiquement pour les journalistes, pour garantir l'exercice de leur mission d'information du public.

pas aux objectifs de la directive de 2019. Concernant les fonctionnaires, la définition proposée ne fait plus mention de la nullité des décisions prises à la suite de discriminations. Il en résultera une prise en compte moindre devant les tribunaux, tant en matière d'annulation de décisions que d'indemnisation. Enfin, le texte proposé restreint par sa rédaction les possibilités de signalement en matière de conflits d'intérêts à un cadre spécifique, impliquant le seul recours au référent hiérarchique ou au référent déontologue. Sur chacun de ces points, cet amendement vise à offrir une nouvelle solution, plus soucieuse de la protection des lanceurs d'alerte et du respect de la directive à transposer.

la commission des lois a entendu clarifier autant que possible cette articulation. Pour ce faire, elle a fait le choix d'inscrire dans la loi Sapin II elle-même la liste des représailles interdites, et d'insérer des renvois à cette liste dans les dispositifs sectoriels. Ce choix de faire de la loi Sapin II le seul texte de référence présente un triple avantage : il renforce la lisibilité du dispositif pour les lanceurs d'alerte eux-mêmes, il évite que certaines catégories de personnes ne demeurent sans protection, et il garantit l'applicabilité des protections prévues contre l'ensemble des mesures de représailles visées par la directive.

plus large, mais qui va dans le même sens.

Pour les raisons que j'ai exposées, le choix de la commission de faire de la loi Sapin II le texte de référence me paraît plus lisible et plus robuste juridiquement. Je vous propose donc de voter l'amendement de la commission plutôt que celui du Gouvernement. La commission émet par

est à Mme le rapporteur. Cet amendement vise à aligner la protection des lanceurs d'alerte militaires sur celle des fonctionnaires civils, moyennant des aménagements rendus nécessaires par la spécificité du statut des militaires.

valeur ajoutée pour les salariés. Si l'on se met à la place d'un lanceur d'alerte potentiel, ce n'est pas dans le règlement intérieur de son entreprise, souvent volumineux, qu'il aura le réflexe d'aller chercher des informations. Il le fera sur internet, auprès de certains de ses collègues ou de référents présents dans l'entreprise, dans des documents de communication interne voire

dès lors qu'ils sont reconnus comme tels. Il a pour objet d'inclure une disposition dans le code du travail afin de permettre aux lanceurs d'alerte de disposer

Premièrement, le lien entre les lanceurs d'alerte, les absences pour formation et les projets de transition professionnelle me semble assez ténu. Deuxièmement, l'avis rendu par le Défenseur des droits vise à donner une première indication à l'auteur d'une alerte sur le respect des conditions de fond et de forme fixées par la loi Sapin mais il n'équivaut en aucun cas à une reconnaissance de la qualité de lanceur d'alerte. Conditionner l'octroi de protections à cet avis ne serait donc pas pertinent et pourrait même induire en erreur quant à sa portée réelle.

qui, eux, sont tributaires des procédures d'urgence de droit commun. Le système serait ainsi beaucoup plus protecteur et permettrait d'appliquer les spécificités de l'alerte à tous, y compris aux agents du secteur public.

La recevabilité du recours en référé-suspension suppose que la décision dont la suspension est demandée n'ait pas été pleinement exécutée. Un lanceur d'alerte particulièrement avisé- qu'il soit agent contractuel de la fonction publique ou fonctionnaire -aura le réflexe de contester son licenciement ou son changement d'affectation la notification de la décision autorisant ceux-ci. Cependant, dans la pratique, accablé par cette procédure de sanction déguisée ainsi que par un contexte de harcèlement ou de pression, le lanceur d'alerte peut effectivement décider d'engager une procédure contentieuse à l'issue de la décision de son licenciement ou de son changement d'affectation, soit quand celles-ci sont pleinement exécutées. Par la suite, la voie du référé-suspension, seul moyen de droit lui permettant d'obtenir une décision protectrice, certes temporaire, mais rapide, lui est fermée.

de la commission ? Ces quatre amendements tendent à rétablir la création d'un référé-liberté « droit d'alerte », où la condition d'urgence serait présumée. La commission a suivi l'avis du Conseil d'État, qui y est franchement défavorable. En l'état, les conditions de mise en oeuvre du référé-liberté permettent au juge administratif de répondre efficacement aux recours des lanceurs d'alerte. Il convient de ne pas complexifier outre mesure le paysage procédural procédural et de ne pas créer une rupture d'égalité entre les requérants, selon la liberté fondamentale dont la violation serait alléguée. Les lanceurs d'alerte disposent, de plus, d'autres instruments procéduraux pour faire valoir leurs droits

ce titre, il tend à consolider le dispositif de l'amende civile prévu par le texte, en supprimant la référence au montant de la demande de dommages et intérêts, en couvrant les procédures civiles et pénales et en unifiant le montant de l'amende à un seuil élevé de 60 000 euros. Quel de la commission ? Cet amendement vise à modifier les modalités du calcul de l'amende civile pouvant être prononcée envers les auteurs de procédures bâillons. Il a pour objet de fixer son montant à 60 000 euros et d'assurer son articulation avec les dispositifs existants dans les codes de procédure civile et pénale.

peine complémentaire dans le code pénal afin de dissuader les entreprises et les organisations qui seraient tentées d'exercer des représailles à l'égard des lanceurs d'alerte. Quel Quel est l'avis de la commission ? L'amendement n° 88 du Gouvernement tend à modifier l'incrimination de la prise de représailles à l'égard d'un lanceur d'alerte. Plutôt que de créer une incrimination spécifique, il vise à rendre applicables aux auteurs de représailles les dispositions du code pénal sanctionnant les auteurs de discriminations. Il renforce ainsi la robustesse juridique du dispositif et assure sa pleine conformité au principe de légalité criminelle. La commission émet donc un avis favorable

La proposition de loi comprend toutefois déjà des sanctions pénales de portée générale à leur endroit et prévoit, en outre, une possibilité de publication des jugements de condamnation. Cet arsenal me semble suffisant, d'autant que le lien entre la peine d'exclusion des marchés publics et la prise de représailles envers un lanceur d'alerte est peu évident. Il me semble

lorsque la procédure engagée est dilatoire ou abusive, et que cela est établi, que le juge puisse condamner l'auteur des faits au paiement d'une amende civile dont le montant serait limité.

permet l'audition sous X des témoins dans les procédures portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition de ces personnes est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. On n'en est tout de même pas

auraient lancée. Il est vrai que le juge dispose déjà de marges de manoeuvre significatives sur ce sujet ; je ne m'oppose donc pas au retrait de cette disposition. Le I de l'amendement soulève en revanche plus de difficultés. L'insertion de nouvelles coordinations dans l'article correspondant du code de justice administrative n'est pas conforme à la démarche de la commission et crée une complexité superflue. Afin de protéger tous les lanceurs d'alerte sans exception, la commission a fait de la loi Sapin II le texte de référence en matière de droit d'alerte et a renvoyé vers celle-ci tous les dispositifs sectoriels. C'est pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement de coordination avec cette logique générale,

divergences de point de vue non négligeables avec la version adoptée par la commission, mais il faut reconnaître que le débat démocratique et constructif auquel nous avons assisté cet après-midi est venu résoudre certains points de désaccord. Ces divergences portaient sur la définition des lanceurs d'alerte, la suppression de la possibilité pour les personnes morales à but non lucratif d'être protégées comme facilitateurs, mais également le champ de l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte et le régime de la divulgation publique. En séance, la mobilisation de plusieurs groupes, l'écoute et l'évolution utile du positionnement de Mme la rapporteure par rapport à celui qu'elle avait eu en commission nous ont permis de dépasser deux de ces difficultés. Nous espérons sincèrement que cet esprit de convergence persistera en commission mixte paritaire, afin que les personnes morales à but non lucratif qui s'exposent en aidant les lanceurs d'alerte puissent être effectivement protégées ou qu'un dispositif cohérent et sécurisant soit trouvé en matière de divulgation publique. L'enjeu est bien sûr d'atteindre l'objectif de renforcer la

vote. Il est plaisant d'observer que notre société cherche à défendre ouvertement ceux qui suivent leur conscience pour que cessent de mauvaises pratiques ou des infractions. Il est parfois nécessaire de braver certaines interdictions pour faire éclater la vérité, pour faire respecter la loi, ou pour la faire évoluer. Je souhaite saluer toutes celles et tous ceux qui se sont engagés avec courage dans cette voie.

Le scrutin est clos. Le scrutin est clos.

Il reviendra au pouvoir réglementaire de le préciser. Sur des affaires particulièrement délicates touchant à des domaines étrangers à ceux qui sont visés par la directive européenne, il pourrait être opportun de laisser plus de six mois à l'autorité externe, plutôt que de lui imposer de fournir une réponse insatisfaisante dans ce délai.

Dans un premier temps, la commission a proposé que le Défenseur des droits soit secondé par un adjoint spécialisé dans ce domaine : il s'agit de répondre de manière pragmatique à une demande formulée par la Défenseure des droits elle-même. Nous verrons ultérieurement s'il y a lieu de

la commission, l'ensemble de la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

a demandé le retour à la procédure normale sur la proposition de loi tendant à expérimenter un chèque emploi petites communes pour l'emploi d'agents contractuels et vacataires inscrite à l'ordre du jour du mardi 1 février prochain. Acte est donné de cette demande. La commission des affaires sociales se réunissant pour établir son rapport et son texte mercredi 26 janvier matin, nous pourrions fixer le délai limite de dépôt d'amendements de séance sur ce texte au lundi 31 janvier à 12 heures. Dans la discussion générale, le temps attribué aux orateurs des groupes serait de quarante-cinq minutes. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé.